Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, au nom de toutes mes collègues présentes dans cet hémicycle, en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je suis très heureuse de présider cette séance de questions d'actualité au Gouvernement. C'est un beau symbole, et je tiens à en remercier sincèrement notre président, Gérard Larcher. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3, sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook.

remercie, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. En cette Journée internationale des droits des femmes, je souhaite évoquer la question des moyens mis en oeuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans son discours du 25 novembre 2017, le chef de l'État déclarait vouloir faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Il s'engageait alors à donner la priorité à la lutte contre les violences faites aux femmes et annonçait une hausse de 13 % des crédits qui On peut s'en étonner, mais en fait de politique publique, celle-là repose essentiellement sur le travail des associations et sur le dévouement de leurs bénévoles. Ces associations remplissent des missions de service public. Or force est de constater que les financements qui leur sont alloués sont non pérennes et souvent insuffisants au regard de l'ampleur des besoins. La libération de la parole a suscité une forte attente, avec un nombre croissant de plaintes de victimes à traiter. Chaque femme est en droit d'attendre un traitement identique de sa plainte, qu'elle habite en ville, dans des territoires ruraux ou d'outre-mer. Or comment mener une vraie politique publique en s'appuyant sur des subventions à la fois incertaines et à géométrie variable selon les territoires ? d'État, en cette journée du 8 mars, pouvez-vous détailler les clés des financements attribués aux violences faites aux femmes ? N'oublions pas que derrière chaque femme victime de violence, il y a également des familles et des enfants victimes.

social Européen. Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la garde des sceaux, nous savons tous que la Protection judiciaire de la jeunesse exerce une mission essentielle, dans des conditions difficiles, pour prendre en charge les mineurs délinquants et les aider à se reconstruire et à s'insérer dans la société. parfois aussi à la société de donner un accompagnement plus personnalisé à ces jeunes, y compris en les plaçant dans des centres éducatifs fermés afin de mieux prévenir la récidive et de les intégrer dans un parcours éducatif. En la matière, des progrès restent à faire pour mieux prendre en compte les spécificités de la délinquance des jeunes filles mineures. Il n'existe en France qu'un seul centre éducatif fermé réservé aux adolescentes, or la mixité peut être véritablement problématique, alors que cette période de la vie est déterminante pour la construction du futur adulte. Ainsi, trop souvent, ces jeunes filles sont placées dans des établissements pénitentiaires pour femmes qui ne répondent pas à leurs besoins spécifiques, malgré le dévouement et le travail remarquable des personnels. Madame la garde des sceaux, les besoins sont réels, vous le savez, mais il nous faut une volonté politique. Ma question est donc simple : envisagez-vous d'orienter, de développer la création de centres éducatifs fermés adaptés aux jeunes filles mineures ? Sachez que, dans tous les cas, en tant qu'élue du Cantal, je suis prête à travailler avec vous pour accueillir une telle implantation sur mon territoire et donner une nouvelle chance à ces jeunes femmes. La parole Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Josiane Costes, les centres éducatifs fermés, qui ont été créés en 2002, sont aujourd'hui au nombre de cinquante-deux sur le territoire national. Ils constituent, vous le savez, une alternative à l'incarcération. Ils permettent d'apporter une réponse « contenante » pour les mineurs qui sont les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves. Ils répondent ainsi à la fois à une forte demande sociale de contrôle et de sécurité, et leur pertinence en matière de prévention

nouveaux centres éducatifs fermés, et il est actuellement envisagé que l'un d'entre eux soit dédié à la prise en charge des jeunes filles. Il n'existe en effet aujourd'hui qu'un seul centre éducatif fermé dédié à des jeunes filles ; il se situe à Doudeville, dans le département de la Seine-Maritime. En 2016, les centres éducatifs fermés, il faut le souligner, n'accueillaient que 6 % de filles, contre donc 94 % de garçons. La perspective dans laquelle nous nous situons répondra au moins pour partie à cette problématique. que la mixité n'est pas un handicap et que, si elle est bien régulée, elle peut être une solution tout à fait satisfaisante. Nous ne savons pas, au moment où je vous parle, quelles seront exactement les localisations choisies pour implanter ces nouveaux centres éducatifs fermés,

Madame la présidente, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la Journée internationale des droits des femmes rappelle chaque année l'actualité de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce 8 mars 2018 restera marqué par la mise au grand jour, salutaire, des violences faites aux femmes dans les sphères privée ou publique. La parole enfin libérée montre que nous ne sommes pas, hélas !, dans le domaine de l'exception. C'est particulièrement vrai sur les lieux de travail. Une femme sur cinq y est victime de violences sexistes ou sexuelles. S'il y a bien obligation pour l'employeur d'agir, de prévenir et de sanctionner, la réalité, froide et cruelle, est tout autre. Nous savons aussi qu'il ne peut y avoir de recul du harcèlement sans recul des inégalités économiques et sociales. Les femmes les plus menacées sont parmi les plus précaires, les plus isolées. Questions sociales et émancipation féminine sont totalement liées. La très grande majorité des femmes font partie des minima sociaux. Elles sont aussi les premières victimes des temps partiels imposés. Et que dire des insupportables inégalités salariales ?

grave encore, ces inégalités salariales entraîneraient un manque à gagner estimé à 246 milliards d'euros de pertes en revenus et cotisations de toutes sortes. De quoi remettre en cause très fortement les vieilles croyances, inspirant les vieilles politiques selon lesquelles le progrès social serait néfaste au progrès économique. C'est tout l'inverse ! L'égalité entre les hommes et les femmes est la grande cause nationale du quinquennat ? Très bien ! Mais, au-delà des effets d'annonce, quels moyens humains et financiers allez-vous mettre en oeuvre ? La

vous avez évoqué deux sujets essentiels en matière de droits des femmes : les violences sexuelles et sexuées au travail et l'égalité salariale. En ce qui concerne les violences sexistes et sexuées au travail,

dans les six à sept semaines qui viennent, afin d'aboutir à des propositions. Ces dernières porteront notamment sur l'information, la formation, la création de référent et les sanctions. Pourquoi la formation ? Parce qu'il est très important que les élus du personnel, les responsables des ressources humaines, les médecins du travail ainsi que l'ensemble des acteurs de la vie de l'entreprise

que lorsque l'on s'attaque au sujet et que l'on progresse en matière de mixité, l'entreprise est plus performante. Il faut donc régler ce problème, d'abord pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons économiques. Avec les partenaires sociaux, nous allons travailler très étroitement sur ce sujet dans les semaines qui viennent.

socialiste et républicain. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre du travail. Madame la ministre, l'égalité est un droit, et c'est bien ce droit que des milliers de Françaises réclament encore aujourd'hui en cette Journée internationale pour le droit des femmes. Lundi, vous annonciez aux Françaises et aux Français un de la formation professionnelle. Trois jours plus tard, vous présentez un plan ambitieux pour lutter contre les inégalités salariales et professionnelles, tandis que, dans le même temps, le Président de la République fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale du quinquennat. Depuis neuf mois, et en toutes matières, les réformes succèdent aux annonces et les projets aux déclarations, avec l'idée affirmée que tout serait à faire et que rien n'a été fait. Ce passé, quel est-il ? Celui d'un ministère de plein exercice,

Quel progrès pour l'égalité des femmes ! Cette égalité, vous le savez, madame la ministre, existe encore moins qu'ailleurs lorsque l'on s'intéresse à la rémunération du travail salarié. Selon votre propre ministère, l'écart moyen entre les salaires des femmes et les hommes s'élève en France à 25,7 tous temps de travail confondus, et à 9 % à poste et expérience équivalents. Alors que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, elles occupent ensuite des postes à moindre responsabilité. En raison des inégalités de carrière, les femmes partent à la retraite un an plus tard que les hommes, avec des droits moins importants. Cette situation est pourtant illégale, parce qu'elle procède d'une discrimination liée au sexe interdite depuis 1982, et parce qu'elle contrevient au principe « à travail égal, salaire égal » prévu par le code du travail depuis quarante-six ans. Quelles mesures entendez-vous prendre pour assurer réellement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ? Pourquoi attendre 2022 pour les mettre en place ? En Islande, la contrainte législative a été immédiate. Quels financements allez-vous pouvoir consacrer aux mesures nécessaires à à la réalité de cette égalité ? J'ajoute, madame la ministre, qu'il est bientôt quinze heures quarante, heure à laquelle les femmes cessent d'être payées chaque jour

la libération de la parole des femmes que nous vivons actuellement et les nouvelles mesures que vous allez mettre en place pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes donnent à cette journée du 8 mars un retentissement tout particulier dont nous ne pouvons que nous féliciter. Mais il est un phénomène qui reste peu connu, mal combattu et particulièrement choquant, je veux parler de la prostitution des adolescentes. Mon intervention repose sur un constat inquiétant, réalisé récemment en Seine-et-Marne : la recrudescence de cas signalés par les forces de police, dont j'imagine qu'il s'agit non pas de cas isolés mais d'une réalité nationale. Des milliers d'adolescentes se prostituent en France dès le collège selon l'association Agir contre la prostitution des enfants, Les profils sont multiples : la réponse à un besoin vital de se nourrir, de payer ses études, le fait de jeunes qui s'y adonnent « parce que ça se fait ». Ce sont principalement des jeunes filles de treize à dix-sept ans, fragiles et souvent déscolarisées.

et les répercussions psychologiques dans leur vie future seront dramatiques. Ne nous y trompons pas, c'est bien de protection des mineures et de dignité humaine qu'il s'agit. Il n'est pas acceptable que, dans notre pays, des jeunes n'aient pas été mieux protégées, mieux orientées, mieux identifiées. Certes, le législateur a fortement investi le domaine de la lutte contre la prostitution des mineurs en instaurant un véritable arsenal répressif, mais la répression ne suffit pas. Aussi, madame la secrétaire d'État, je vous demande de lancer une étude d'envergure pour connaître plus précisément l'ampleur du phénomène, préalable indispensable à la mise en place de mesures de sensibilisation, de prévention, de formation tant des travailleurs sociaux, ... Veuillez conclure,

Enfin, je voudrais ajouter que ces sujets, et particulièrement celui de la prostitution des mineurs que vous évoquez, s'inscrivent pleinement dans le plan de protection de l'enfance qui sera présenté dans le courant de 2019 par ma collègue ministre des solidarités et de la santé. Vous le voyez donc, tout le Gouvernement est mobilisé sur cette question cruciale.

Républicains. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame la secrétaire d'État, cela fait plus de quarante ans que des lois imposent comme principe essentiel l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Or, en 2018, l'écart salarial à poste égal est de 10 %. C'est une différence injustifiée et une véritable discrimination. Et c'est un échec collectif, vous venez

Mais l'exemple doit venir du sommet de l'État. Vous avez récemment déclaré, madame la secrétaire d'État, que, dans le monde professionnel, lorsqu'on cherche des femmes compétentes, on en trouve. Pourriez-vous donc être notre porte-parole auprès du Président de la République, car, parmi les douze conseillers nommés auprès de lui, on ne compte qu'une seule femme

C'est la Journée internationale des droits des femmes ! ... je veux appeler votre attention sur une population souvent oubliée et parfois abandonnée : les femmes incarcérées. Au 1 janvier 2018, nous en comptions près de 3 000. Dans un premier temps, je tiens à saluer la décision visant à installer, au mois de septembre prochain, une crèche pour accueillir les bébés à Fleury-Mérogis. Cette mesure de bon sens mérite d'être généralisée. Cependant, comme un arbre qui cache la forêt, cette bonne nouvelle masque une situation plus contrastée. Les défis à relever sont encore immenses, en particulier pour ce qui concerne les conditions de détention En effet, dans certains établissements, notamment à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, un accès limité et non quotidien aux douches est à déplorer, tandis que les hommes ont des douches à leur disposition dans leur cellule. Cette triste réalité conduit le personnel soignant à prescrire des « douches médicales ». Cette inégalité de fait est inacceptable. Par ailleurs, d'autres difficultés sont à souligner les faibles activités proposées, qui sont souvent limitées aux seules activités ménagères ; la localisation géographique des établissements, complexifiant ainsi le maintien des liens familiaux ; sans oublier l'accès aux soins, notamment les soins gynécologiques. Comme l'a si bien rappelé la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans son avis du 25 janvier 2016, « le principe d'égalité entre les hommes et les femmes doit s'appliquer dans l'intégralité de la société, celle du " dehors " comme celle du " dedans ", et les personnes privées de liberté doivent également en bénéficier sans restriction

». Mais je pense plus précisément à elle parce qu'elle a également explicité dans cette même déclaration que la rigueur de la loi pénale devait s'appliquer de la même manière aux hommes et aux femmes ; c'est une autre version du principe d'égalité. Or la question que vous soulevez a précisément à voir avec ce principe d'égalité.

la dignité, le suivi du parcours de détention et la sécurité, bien sûr, pour la société, comme à tout détenu. Nous héritons d'une situation que nous devons prendre en charge et à laquelle nous devons bien entendu trouver des réponses. Cette situation est de nature immobilière. Vous l'avez relevé, à juste titre, les quartiers des femmes sont souvent situés dans des endroits vétustes-

Ma question s'adresse à M. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Une commission indépendante composée d'experts, mandatée par le Premier ministre et présidée par l'économiste Katheline Schubert, a remis, en septembre dernier, au Gouvernement un rapport l'alertant sur les impacts environnementaux, climatiques et sanitaires de l'Accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA. Confirmant en partie les craintes qui s'étaient exprimées, les rapporteurs ont fait preuve d'inventivité en proposant la création d'un « veto climatique » face aux impacts de certaines dispositions envisagées quand les objectifs en matière de respect des enjeux liés au développement durable et des accords climatiques ne sont pas respectés et sont « loin d'être atteints ». À la suite de ces recommandations, vous avez, monsieur le ministre d'État, intégré le principe du veto climatique dans le plan d'action du Gouvernement sur le CETA, sans toutefois en donner les conditions juridiques d'opérationnalité, ce qui a entraîné le scepticisme des ONG environnementales. Aujourd'hui, les discussions sur les échanges commerciaux avec l'Amérique latine sont en cours dans le cadre du Mercosur. De nombreuses questions de compatibilité des modes de production et de consommation entre les parties prenantes sont là encore au coeur des débats, notamment concernant l'agriculture, et plus particulièrement l'élevage bovin. Le groupe radical du Sénat a d'ailleurs déposé une proposition de résolution, portée par le président Requier, sur ce volet. Nous pouvons aussi aisément ajouter aux impacts sur l'économie de la viande bovine en France et en Europe les conséquences en termes climatiques, puisque cette production est, nous le savons, fortement émettrice de gaz à effet de serre et responsable de déforestation. Monsieur le ministre d'État, nous partageons, me semble-t-il, la conviction que les négociations commerciales sont un des principaux leviers de mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat. Je souhaite donc vous poser une double question. Premièrement, avez-vous défini les critères d'instauration du veto climatique,

La parole est à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Ronan Dantec, je rêve d'un temps que j'espère proche où l'on parlera non plus d'accord ou de traité de libre-échange, mais d'accord ou de traité de juste échange. Vous m'interrogez, monsieur le sénateur, à juste titre- vous savez que je partage votre préoccupation -sur la mise en oeuvre du veto climatique dans le cadre du CETA

cela prendrait la forme d'une nouvelle déclaration juridique interprétative, qui devrait être adossée à la partie consacrée aux investissements du CETA, mais il nous faut encore obtenir l'accord du Conseil avant de pouvoir finaliser le dispositif avec le Canada. Je ne vous le cache pas, nous devrons faire durant le printemps un véritable travail de conviction à la fois auprès de nos partenaires européens et évidemment de nos amis canadiens. S'agissant du Mercosur, vous avez probablement entendu le Président de la République déclarer très clairement devant les jeunes agriculteurs le 22 février dernier : il y a des lignes rouges en matière d'indications géographiques, sanitaire et phytosanitaire, mais aussi de respect de l'accord de Paris. C'est bien parce que ces lignes rouges ont été affirmées que l'accord n'a pas encore été conclu. Le Président de la République avait alors aussi rappelé que l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur n'entrerait pas en vigueur tant que l'Union n'aura pas renforcé ses normes sanitaires et environnementales et que l'on n'aura pas obtenu de garanties quant au respect de ces normes. La France s'opposera à la mise en oeuvre du Mercosur si ce travail n'est pas fait en amont. L'accord n'entrera donc pas en vigueur si nous n'avons pas satisfaction sur ce point. La

la formation professionnelle est la pierre angulaire de la lutte contre le chômage et du renforcement de la compétitivité des entreprises. La volonté, louable, de réformer la formation professionnelle n'est pas nouvelle : l'atteste la création du compte personnel de formation, le CPF, sous le précédent gouvernement. Votre projet contient certaines avancées pour les travailleurs, j'en conviens : droit à la formation accru pour les salariés faiblement qualifiés, création d'un compte personnel de formation de transition, par exemple. Mais il est aussi porteur d'interrogations, d'inquiétudes, de défiance, de regrets. D'abord, sur la méthode d'un big-bang, au moins pour le volet gouvernance, proposé de manière unilatérale, sans concertation, sont nées, au premier rang desquelles la monétisation du CPF. Comment ne pas craindre un affaiblissement du droit à la formation de certains salariés ? Les 500 euros d'aujourd'hui ou de demain suffiront-ils à financer les 20 heures de formation d'hier, et ce dans tous les territoires ? nous interrogeons sur la place des régions dans la gouvernance de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Votre projet opère un transfert des organismes organisme ne doit pas conduire à écarter les branches professionnelles ni les organisations syndicales de la définition des besoins en compétence. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point ? La réforme, enfin, va dans le sens de l'individualisation. Mais la formation professionnelle ne peut se réduire à « un clic » une application mobile. Ces éléments ne doivent pas entraîner une régression de l'accompagnement du salarié dans l'exercice de son droit à la formation. Madame la ministre, le big-bang annoncé sera-t-il à la hauteur des attentes sociales et des mutations de notre économie Le doute est permis quand ni les chômeurs de longue durée, ni les travailleurs handicapés, ni les indépendants n'y ont trouvé place. La parole

les ouvriers et les employés ont deux fois moins de chances de se former que les cadres, alors qu'ils n'ont pas moins de besoins ; seul un chômeur sur dix a accès à la formation chaque année

professionnelle, nous ferons le même constat sur le plan social : le train de la croissance va reprendre, entraînant des créations d'emplois, et une grande partie de nos concitoyens ne pourront pas monter dans ce train parce qu'ils n'auront pas les compétences nécessaires.

Depuis dimanche dernier, l'Italie observe au Palais du Quirinal le président Sergio Mattarella tenter de dénouer le noeud gordien issu des urnes ... Tout comme la France observait il y a soixante ans le président René Coty à l'Élysée. C'était chez nous le temps de la proportionnelle avec ses majorités éphémères, construites sur des compromis de couloir. C'était le temps où l'on changeait de gouvernement tous les cinq mois. Aujourd'hui encore, il y a des pays sans exécutif, avec un gouvernement sortant qui expédie les affaires courantes.

Car, au-delà des formes multiples que prennent, dans chaque pays, les expressions extrêmes ou démagogiques, il existe, monsieur le Premier ministre, un dénominateur commun à tous ces exemples la proportionnelle intégrale ou partielle. Grâce au général de Gaulle et aux pères fondateurs de la V République, les Français élisent, quant à eux, leurs députés au scrutin majoritaire à deux tours. Ils bénéficient en retour de majorités claires et stables. Monsieur le Premier ministre, au vu des situations vécues par nos voisins et amis, le Gouvernement est-il toujours enclin à introduire une dose substantielle de proportionnelle ? Peut-il prendre le risque d'ajouter à terme aux difficultés économiques du pays une crise politique ?

Le débat entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel est ancien. Je me permets de vous faire observer, monsieur le sénateur, que la V République elle-même a vécu pendant un temps avec un scrutin proportionnel intégral.. Merci Mitterrand ! Si l'on peut s'interroger sur ! Si l'on peut s'interroger sur les décisions qui ont été prises par les majorités issues de ces scrutins, personne, monsieur le sénateur- et certainement pas le Sénat ! -, aucun citoyen de bonne foi ne peut dire que les institutions auraient été pendant ces années-là bloquées. En aucune façon

que ce qu'elles donnent à voir. Je me permets enfin de vous faire remarquer que le système allemand, qui repose sur la proportionnelle, a permis le renouvellement pendant plusieurs mandats des mêmes majorités,

Si je vous dis cela, monsieur le sénateur, c'est parce que le Président de la République s'est engagé pendant sa campagne à introduire une dose de proportionnelle dans la désignation des députés. Je relève d'ailleurs que la dose de proportionnelle existe au Sénat, et je n'ai pas compris que vous proposiez de revenir sur une dose de proportionnelle pour l'élection des députés ? Pour permettre à des pans assez larges de la population française et des électeurs français d'avoir la garantie d'être représentés

Vous avez parfaitement le droit de le penser ! Je ne pense pas que l'introduction de 10 %, 15 %, 20 % ou 25 % de proportionnelle soit de nature à remettre en cause les institutions ; en témoigne la proportionnelle intégrale en 1986, qui n'avait d'ailleurs pas empêché le Sénat de fonctionner.

La V République a assuré la stabilité politique en France. C'est l'un des legs les plus précieux du général de Gaulle. Revenir au scrutin proportionnel, c'est le retour au vieux monde, celui de l'instabilité politique, celui des tractations entre appareils politiciens comme « au bon vieux temps » du régime des partis. Le scrutin majoritaire est indissociable de la logique de nos institutions. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour le groupe Les Républicains.

universitaire de Saint-Étienne, du 8 au 15 janvier 2018, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées dans cet établissement. Elle a observé des conditions d'accueil indignes au sein du service des urgences générales, des pratiques abusives d'isolement et de contention dans les unités d'hospitalisation complète, ainsi qu'un défaut d'information des patients sur leurs droits. La Contrôleur déplore que « les conditions de vie de certaines personnes hospitalisées constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme Cette situation s'explique par le manque de places d'hospitalisation dans les services de psychiatrie. Elle n'est pas exceptionnelle, mais plutôt symptomatique des difficultés qui touchent la psychiatrie en France. Elle est la conséquence de plusieurs paramètres bien identifiés : la baisse des moyens alloués aux services de psychiatrie et le problème de la formation. En trente ans, le nombre de lits dans ces services a été divisé par deux. Mille postes de psychiatres restent vacants, et la spécialité d'infirmier psychiatrique a disparu depuis les années Conformément à la loi, Mme la ministre des solidarités et de la santé a été destinataire de ces recommandations. Un délai de trois semaines a été donné pour y répondre. Or, à l'issue de ce délai, aucune réponse de l'autorité compétente n'est parvenue.

l'un des combats majeurs de notre organisation nationale de santé. Elle assurera personnellement la présidence de l'instance nationale, le comité stratégique de psychiatrie et de santé mentale.

la psychiatrie est inscrite comme l'une des thématiques prioritaires du programme hospitalier de recherche clinique pour 2018. Il est évident que la recherche française doit être accompagnée, afin de continuer à progresser sur ce sujet. En même temps, il faut que nous trouvions des réponses territorialement adaptées

Le rayonnement de la France dans le monde passe par nos écoles, nos collèges, nos lycées français à l'étranger. Or votre gouvernement procède à des coupes claires et d'une violence inouïe à l'encontre de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, qui concerne 495 établissements scolaires répartis dans 137 pays et scolarise 342 000 élèves dans le monde. En effet, en coupant de 33 millions d'euros, c'est-à-dire 10 % du budget de l'Agence, brutalement, sans concertation, sans méthode, vous fragilisez, vous mettez en danger l'avenir de nos écoles françaises à l'étranger, et ce pour plusieurs raisons.

ou bien allez-vous changer de politique et faire ce qu'il conviendrait de faire, c'est-à-dire vous battre pour nos écoles et nos lycées français à l'étranger, qui sont le fer de lance de la francophonie, qui incarnent la voix de la France dans le monde et qui, d'une certaine manière, à l'image de ce que disait le général de Gaulle, incarnent « une certaine idée de la France » ? La parole

Il assure deux missions : une mission de service public pour les enfants de nos compatriotes installés à l'étranger et une mission d'influence puisque deux tiers des enfants qui y sont scolarisés sont étrangers. En termes budgétaires, c'est la première priorité de notre diplomatie d'influence, avec 60 % du programme 185, et cela va le demeurer. ! Oui, en 2017, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a fortement contribué aux annulations de crédits rendues nécessaires par l'état de nos finances publiques. Au total, 282 millions d'euros ont été annulés, dont 33 millions d'euros, c'est vrai, ont porté sur l'AEFE. Dans ce contexte, j'entends comme vous les inquiétudes exprimées, mais je voudrais vous rassurer. Je rappelle d'abord l'engagement du Président de la République, qui a salué devant l'Assemblée des Français de l'étranger le travail de l'AEFE et de ses personnels. Il a confirmé que ses crédits seraient préservés en 2018 et en 2019. J'ajoute qu'une dotation exceptionnelle de 14 millions d'euros a été ajoutée pour des questions de sécurité. de sécurité. J'indique également que le Président de la République a demandé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui présenter, en lien avec le ministre de l'éducation nationale, des propositions à l'été pour réformer l'Agence. La situation budgétaire de celle-ci l'exige, afin de pouvoir consolider le modèle des lycées français à l'étranger, auquel nous sommes profondément attachés. Les moyens d'abord ! Cette stabilité budgétaire doit permettre de conforter l'AEFE dans la durée, sur la base d'une stratégie à la hauteur des deux grands défis que rencontre notre réseau

En Marche. Monsieur le Premier ministre, voilà plus de trois semaines que la population de Mayotte, lasse des violences au quotidien, manifeste contre l'insécurité, bloque les routes. Les fonctionnaires et les transporteurs exercent leur droit de retrait. Les services municipaux et départementaux sont fermés, en solidarité. La journée d'hier a été marquée par une forte mobilisation populaire. Il ne s'agit pas seulement des caillassages dont sont victimes les lycéens, des agressions sur les routes, dans les villages et les maisons, ni de l'insuffisance de la réponse pénale. Les violences, c'est aussi l'embolie du système éducatif ; ce sont, dans un contexte de forte pression migratoire, les difficultés considérables d'accès aux soins, le manque de logements décents, la faiblesse des infrastructures, l'absence des services et de l'encadrement qui existent partout ailleurs en France. La maternité de Mamoudzou est celle qui enregistre le plus de naissances en France. Quel avenir les parents qui ont défilé en si grand nombre hier peuvent-ils offrir à leurs enfants sur un territoire où la moitié de la population a moins de dix-huit ans ? Des premières mesures ont été annoncées, dont le renforcement des forces de l'ordre, la création d'une brigade de prévention de la délinquance juvénile et un plan de sécurisation des établissements et des transports scolaires. Mme la ministre des outre-mer a affirmé avec justesse que la seule réponse sécuritaire ne suffisait plus et propose la tenue d'une conférence pour l'avenir de Mayotte, après les résultats des assises. Vous comprendrez bien que la population ne puisse pas attendre jusque-là, car les besoins sont connus et appellent des mesures urgentes, globales et concrètes. Tiendrez-vous compte des propositions adressées au Président de la République par l'ensemble des forces vives du département, qui appellent unanimement à un plan de développement le groupe La République En Marche et les sénateurs mahorais, en cette journée particulière où, dans mon département, on se souvient de la lutte des chatouilleuses pour le choix de la France, vous le demandent solennellement : que répondez-vous à ceux qui pensent que la République a abandonné Mayotte ?

ils sont inquiets pour leur sécurité, en premier lieu pour celle de leurs enfants, pour la sécurité dans les écoles. Ils attendent des réponses.

Toutes les dispositions ont été prises pour qu'aucun élève, aucun enseignant ni aucun agent travaillant dans les établissements ne soit menacé trois escadrons de gendarmerie mobile sont en cours de déploiement sur l'île, ainsi que des agents de sécurité et des médiateurs de l'éducation nationale ; des forces supplémentaires arriveront mardi. Avec Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur, nous avons prévu une mobilisation totale des forces de l'ordre. Cela n'est toutefois pas suffisant- vous avez raison. Il faut aller plus loin, car nos compatriotes attendent des réponses à la fois urgentes et rapides en matière de sécurité, mais aussi de lutte contre l'immigration clandestine, de santé, de logement et de transport. Des réponses rapides et urgentes, monsieur le sénateur, à des problèmes qui ne sont pas récents.

en 2002, 160 000, en 2007, 186 000 et en 2012, 212 000

simplement, je crois utile de rappeler que le mécontentement qui s'exprime aujourd'hui, et qui doit être entendu, parce qu'il est légitime, ne naît pas d'une situation récente, mais de la construction d'une situation qui

sur l'organisation institutionnelle et l'organisation des politiques publiques qui permettent de définir des solutions. Nous voyons bien la question, que vous avez mentionnée, de la maternité, qui enregistre plus de 10 000 naissances par an, soit deux fois plus que la plus grande maternité parisienne. Comment traiter cette question ? Doit-on s'autoriser à travailler sur un nouveau statut de cette maternité ? Réfléchir aux transformations qu'il faudrait opérer en matière de droit et d'accès à la nationalité à cet endroit ? Je mets tout sur la table, monsieur le sénateur, mais je veux dire que les appels au « décasage », non plus que les barrières ou les barrages qui seraient installés sur les routes, n'apporteront rien aux habitants de Mayotte : ils ne permettront rien

eux. Il nous faudra formuler des propositions en assumant les difficultés spécifiques auxquelles est confronté ce cent unième département français.

Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au Gouvernement auront lieu le mardi 13 mars, à seize heures quarante-cinq ; elles seront retransmises sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat, ainsi que sur Facebook.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque, en 2013, j'ai présenté mon rapport sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, devenu la loi du 2 janvier 2014, j'ai indiqué que de nombreuses suggestions complémentaires de simplification ou de clarification m'avaient été présentées lors de mes auditions. Compte tenu des délais d'examen de ce texte et de sa composition à base, pour l'essentiel, j'avais préféré renvoyer l'examen de ces suggestions à un travail complémentaire, susceptible de donner lieu à l'élaboration d'une proposition de loi spécifique. Aussi ai-je déposé, le 4 août 2014, la présente proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce. J'ai souhaité passer au crible de l'impératif de simplification, aujourd'hui partagé unanimement, les dispositions du code de commerce laissées de côté, pour formuler dans un texte à l'objet à l'objet clair et circonscrit des simplifications, des clarifications et des mises à jour concrètes objectivement utiles pour la vie économique. La finalité de cette proposition de loi est simple, mais ambitieuse : améliorer la compétitivité de l'économie française et réaliser des économies budgétaires. Il n'était pas question de simplifier pour s'inscrire dans l'air du temps. La complexité de la règle de droit n'est parfois que le reflet de la complexité de la réalité économique. En revanche, lorsque cette complexité n'a pas lieu d'être ou n'a plus de justification dans la réalité, elle n'a pas à être conservée. Pour autant, la simplification ne doit pas méconnaître l'aspiration des acteurs économiques à la stabilité de la règle de droit. Ces deux exigences ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. À la lumière de ces exigences et à l'aide du regard des praticiens, il est possible de simplifier avec mesure et pragmatisme. C'est ainsi que je conçois toute oeuvre de simplification vraiment utile pour nos entreprises. À cet égard, la succession de trains de simplification depuis de nombreuses années a parfois manqué de lisibilité pour les acteurs et les praticiens du droit des entreprises, contraints de prendre en compte de fréquentes modifications des règles applicables. Comme la complexité du droit, l'instabilité normative a un a un coût économique, que les pouvoirs publics doivent prendre en compte et chercher à minimiser. Ainsi, je crois parfois préférable de maintenir une règle complexe ou apparemment lourde, mais comprise et largement acceptée, plutôt que de la changer au profit d'une règle nouvelle certes objectivement plus simple mais qui exigera un effort d'adaptation excessif de la part de tous. J'avais également à coeur que la simplification de l'environnement juridique des entreprises ne s'opère pas au détriment de la protection des intérêts des tiers, salariés, actionnaires, clients et fournisseurs, à laquelle contribue fortement, entre autres dispositifs, la publicité légale. Il est indispensable de préserver un équilibre entre simplification du droit, secret des affaires et protection des intérêts des tiers, comme l'a fait, par exemple, l'ordonnance du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et petites entreprises. Il appartient bien au législateur d'arbitrer entre des mesures de simplification réellement utiles et le besoin de stabilité de l'environnement juridique des entreprises et,, de

Notre droit des entreprises ne doit pas être une cause de délocalisation des activités économiques. Après vous avoir présenté mon objectif, j'en viens à la méthode retenue pour y parvenir. J'ai souhaité circonscrire mon travail au droit des sociétés. Dans ce champ restreint clairement identifié, j'ai fait le choix de partir des besoins exprimés par les acteurs de la vie économique- autorités administratives indépendantes, représentants des entreprises, professionnels accompagnant les entreprises, -pour déterminer des mesures concrètes et utiles de simplification, de clarification ou d'actualisation. Supprimer des obligations obsolètes ou n'atteignant pas leur objectif, alléger des contraintes inutilement lourdes, complexes ou disproportionnées, corriger des erreurs ou des incohérences résultant de la sédimentation de textes successifs, clarifier des dispositions ambiguës posant des difficultés d'interprétation, harmoniser des rédactions disparates, renforcer la sécurité juridique, rendre plus efficaces certains mécanismes conformément à leur finalité, faciliter l'accomplissement de certaines procédures ou formalités, parfois en les dématérialisant, éviter les dispositifs trop rigides ou excessifs au profit de la liberté des parties, fluidifier les relations économiques et la vie des affaires sans remettre en cause la protection des divers intérêts en présence : tels sont les axes que j'ai retenus pour élaborer la proposition de loi. En dépit de ce champ réduit, le présent texte se composait initialement de soixante articles. Après son passage en commission, en 2016, il en comptait toujours de nombreuses mesures ont été reprises dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, et dans la loi du 10 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II. Je tiens d'ailleurs à saluer l'excellent travail de notre rapporteur, André Reichardt, qui a su, à l'époque, enrichir ce texte et qui l'a, aujourd'hui, épuré de toutes les dispositions satisfaites.

ce qui, vous en conviendrez, relève presque du défi. Pour corser encore notre exercice, et parce que je nous sais capables de relever ce défi, j'ai souhaité déposer quatre amendements compléter et à actualiser le travail débuté en 2013. Le premier vise à ratifier quatre ordonnances prises par le Gouvernement en 2017 dans le domaine du droit des sociétés. ont repris plusieurs dispositions de la proposition de loi, dans une rédaction parfois différente, ce qui montre bien, en tout cas, la convergence de vues qui existe en matière de simplification du droit des sociétés. amendement tend à simplifier le dispositif permettant la dématérialisation des assemblées générales d'actionnaires dans les seules sociétés anonymes non cotées, afin de le rendre enfin applicable. La proposition de loi comporte un dispositif en ce sens. L'ordonnance du 4 mai 2017 sur la participation des actionnaires a mis en place un dispositif qui s'en inspire : les statuts de la société peuvent prévoir la tenue de l'assemblée générale de façon dématérialisée, puisque cette faculté relève des statuts, ce sont les actionnaires qui auront à accepter ou non, dans le cadre d'une modification des statuts, une telle faculté. Or l'ordonnance ajoute un droit d'opposition à la tenue dématérialisée de l'assemblée générale pour les actionnaires représentant au moins 5 % du capital, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. À ce jour, le décret n'a toujours pas été pris, alors que l'ordonnance date de mai 2017 Ce dispositif, pourtant attendu par les praticiens du droit des sociétés, n'est donc toujours pas opérationnel. En réalité, ce décret est sans doute très difficile à élaborer pour concevoir les modalités, en particulier chronologiques, du droit d'opposition. Le plus simple est donc de supprimer ce droit d'opposition, dont l'utilité n'est pas avérée dans les sociétés non cotées, dès lors que les actionnaires ont la faculté de s'opposer à la possibilité de réunions dématérialisées au stade de la modification des statuts en assemblée générale extraordinaire, laquelle requiert des niveaux très élevés de quorum et de majorité. a pour objet de simplifier les règles de rachat par une société non cotée de ses propres actions, en ménageant plus de souplesse. L'objectif est simple : favoriser l'entrée d'investisseurs extérieurs destinés à accompagner la croissance de l'entreprise, en particulier en facilitant leur sortie du capital, le moment venu, par le rachat des actions qu'ils détiennent. Il n'existe pas, en effet, de réel marché pour les actions des sociétés non cotées. Lorsqu'une telle opération de rachat est soumise à l'assemblée générale des actionnaires, un rapport du commissaire aux comptes suffit, compte tenu des garanties de déontologie et d'indépendance de ce dernier. Le rapport supplémentaire d'un expert indépendant est redondant et ne donne pas une information supplémentaire utile aux actionnaires. il est bon de prévoir que l'opération de rachat, autorisée par les actionnaires pour une durée limitée, peut être utilisée pour les différentes finalités permises par la loi, et pas seulement pour une finalité donnée. Cette souplesse restera encadrée par la loi. Enfin, les actions de préférence ont été créées en 2004, puis réformées en 2008 et 2014, mais sans rencontrer le succès attendu. Elles restent peu utilisées, alors même

pour rendre celles-ci plus attractives. Certaines sont plus techniques : par exemple, pour les sociétés par actions simplifiées ou pour la suppression du droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital. D'autres ont une plus grande portée, comme la possibilité pour le conseil d'administration de garantir le versement de dividendes à des actionnaires détenteurs d'actions de préférence ou la possibilité de rachat des actions de préférence sur l'initiative de leurs détenteurs à l'issue d'une période donnée, qui n'existe pas aujourd'hui. Comme pour le rachat des actions dans les sociétés non cotées, il s'agit d'encourager l'investissement dans les sociétés en croissance et le capital-risque. C'est indispensable pour la croissance des entreprises françaises. j'ai tenu à conduire cette démarche dans un esprit consensuel, pragmatique et constructif, dans l'intérêt de nos entreprises. C'est la raison pour laquelle j'invite notre assemblée à voter la proposition de loi, pour que ce travail utile pour nos sociétés ne se perde pas dans les méandres de la procédure parlementaire.

limitée à quatre heures. Or j'entends bien, avec votre concours, faire enfin adopter cette proposition de loi, dont le parcours a été pour le moins chaotique,

en 2018, un texte qui sera voté, je l'espère, plus de quatre ans après son dépôt. Un tel parcours, chaotique pour le moins, me paraît regrettable, car le texte comporte, depuis l'origine, un certain nombre de mesures de simplification utiles et attendues par nos entreprises. Je remercie donc le groupe La République En Marche d'en avoir demandé l'inscription à l'ordre du jour du Sénat cet après-midi. Je veux aussi saluer l'inspiration

En dépit des discours répétés en faveur de la simplification et de l'allégement des charges administratives des entreprises, nous nous sommes rendu compte qu'il n'est pas simple de simplifier, compte tenu de la surcharge de l'ordre du jour législatif. Simplifier est un travail ingrat, minutieux, peu visible politiquement et peu prioritaire. Il suffit, mes chers collègues, de voir notre hémicycle ... Le sort réservé à cette proposition de loi jusqu'à présent l'illustre parfaitement. Certes, un certain nombre de dispositions de la proposition de loi ont été reprises par d'autres textes depuis que nous l'avons examinée en commission, en juin 2016, en particulier par la loi du 9 décembre 2016,

Sans m'étendre sur le contenu de la proposition de loi, j'en citerai quelques mesures, toujours d'actualité et très attendues par les entreprises et tous les praticiens : les modalités d'octroi de garanties à une filiale contrôlée, le décompte des abstentions dans les assemblées générales, l'assouplissement des « fenêtres négatives » en matière d'attribution de stock-options et de cession

cette proposition de loi démontre que l'initiative parlementaire authentique- nous nous sommes efforcés qu'elle le soit -peut prendre sa part de l'oeuvre de simplification du droit, secteur par secteur, loin de la méthode fourre-tout de certaines lois de simplification passées dont je ne citerai pas l'auteur, que notre ancien collègue Bernard Saugey avait qualifiées d'« assemblage hétéroclite de cavaliers législatifs en déshérence » ... Comme c'est bien dit ! Dans nos commissions permanentes, mes chers collègues, nous pouvons faire ce travail et passer au crible un pan complet du droit pour en retirer une série de mesures de simplification sectorielles, ciblées et évaluées. C'est ce que M. Mohamed Soilihi a voulu faire, et je m'en félicite. Encore faut-il, bien sûr, que de tels travaux puissent aboutir en séance publique. Tel est le cas cet après-midi, et c'est tant mieux. Dès lors, monsieur le ministre, alors que vous allez bientôt présenter le projet de loi pour un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, nous comptons sur vous- je me permets de compter sur vous -pour que cette excellente initiative puisse suivre son cours

et qui voient les obstacles auxquels ils sont confrontés en termes de complexité juridique savent qu'il faut simplifier le code de commerce. Je tiens à saluer le travail accompli par le rapporteur, André Reichardt

la même idée-force de simplification de la vie des entrepreneurs. Ce sont ces entrepreneurs qui créeront les emplois dont nous avons besoin ; ce sont eux qui créeront les richesses et la prospérité dont nous avons besoin c'est à eux qu'il faut donner les moyens de développer leurs activités pour être concurrentiel par rapport à nos grands voisins et partenaires européens ; c'est à eux qu'il faut répondre quand ils disent que certains obstacles juridiques sont incompréhensibles et les empêchent de développer leur activité dans de bonnes conditions.

c'est parce que nous produirons plus que nous pourrons partager davantage, et c'est parce que nous aurons permis à nos entreprises de grandir que les salariés pourront avoir une meilleure rémunération à la fin du mois. Voilà notre objectif : faire en sorte que les salariés soient mieux récompensés, que le travail soit mieux récompensé,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, rien n'est jamais trop simple dans l'existence. Nul doute que notre collègue Thani Mohamed Soilihi pourrait faire sienne

nous étions face à un texte qui comprenait soixante articles. Un certain temps, et même un temps certain, s'est écoulé entre le dépôt de la proposition de loi et la publication du rapport au fond, à tel point que le texte s'est trouvé amputé d'une bonne vingtaine d'articles avant d'en regagner une douzaine pour les raisons les plus diverses.

dispositions figurant dans cette proposition de loi sont reprises dans la lettre d'articles issus de l'une des ordonnances promulguées dans le courant de l'année 2017 et dans le droit fil de la loi Sapin II. plus précisément de l'ordonnance sur le commissariat aux comptes, issue de la loi Macron : celle-ci a été ratifiée et les articles de la proposition de loi qui y font référence n'ont de fait plus de raison d'être. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 qui a repris les termes de l'article 60 de la proposition de loi sur la question très importante de la responsabilité environnementale des entreprises qui

portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés. On observera dans ce cas qu'il existait en parallèle une proposition de loi en attente d'examen et une ordonnance en instance de ratification qui un objectif similaire. De notre point de vue, si l'on peut apprécier la teneur des articles de l'ordonnance portant sur le document de référence présenté aux actionnaires comme aux instances représentatives du personnel lors des assemblées générales ordinaires pour retracer la vie de l'entreprise sur l'exercice comptable, on ne peut en revanche pas tout à fait souscrire aux articles qui réduisent

toujours pas ratifiée, autorise l'organisation d'assemblées générales par visioconférence et reconnaît, même de façon limitée, le droit aux actionnaires minoritaires de faire porter certaines questions à l'ordre du jour.

un tel traitement de l'initiative parlementaire me paraît justifier que nous nous interrogions sur le sens actuel de la démocratie représentative et les modalités d'exercice du pouvoir comme de la confection de la loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'objectif de simplification de la vie des entreprises, aujourd'hui de plus en plus partagé, peut être atteint par le biais de divers leviers, qu'il s'agisse du droit du travail, du droit fiscal ou du droit social. L'actualisation du code de commerce en fait également partie : de nombreuses contraintes, inutilement lourdes et complexes, pèsent en effet sur les sociétés, auxquelles viennent s'ajouter des obligations parfois ambiguës, incohérentes, voire obsolètes. En conséquence, c'est un sentiment d'insécurité juridique qui prédomine pour une partie des sociétés françaises. Il était donc absolument nécessaire de s'atteler à une clarification et une actualisation de notre code de commerce. Ce vaste chantier de simplification a été ouvert il y a quelques années déjà

puisque la plupart des mesures ont été circonscrites au champ du droit des sociétés. Monsieur Mohamed Soilihi, cher collègue, mettre à profit les travaux que vous aviez précédemment menés en tant que rapporteur de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Les besoins de ces dernières ont été cernés avec acuité, et le travail que vous avez accompli saura sans nul doute combler leurs attentes. Je profite d'ailleurs du temps qui m'est accordé pour saluer l'initiative de nos collègues du groupe La République En Marche, qui ont déposé un amendement visant à ratifier quatre ordonnances prises en en 2017 dans le domaine du droit des sociétés. Dans la mesure où les dispositions de ces ordonnances rejoignent celles de la proposition de loi sur plusieurs points, cette ratification nous paraît tout à fait opportune.

Certaines portent sur les fonds de commerce, et visent à en simplifier les formalités de cession et les conditions de mise en location-gérance. D'autres concernent les commissaires aux comptes et prévoient d'assouplir certaines règles d'incompatibilité ou de secret professionnel. Néanmoins, le coeur du texte a trait à la simplification du droit des sociétés, que ces dernières soient de nature civile ou commerciale. Des incohérences sont supprimées, à l'image de l'impossibilité actuelle d'annuler une décision des associés de SARL- ou société à responsabilité limitée -prise en violation des règles de délibération. Certaines règles de fonctionnement des sociétés sont également assouplies, puisqu'il est question de dématérialiser la tenue des assemblées générales des sociétés anonymes, en utilisant par exemple les outils de visioconférence et de télécommunication. Enfin, certaines procédures lourdes et complexes sont allégées. Je souhaiterais revenir à cet égard sur le contenu de l'article 18, dont les dispositions visent à faciliter les conditions d'octroi de cautions, d'avals et de garanties par une société mère à ses filiales. Rappelons qu'en l'état du droit ces cautions, avals et garanties consentis par des sociétés autres que des sociétés exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent avoir reçu l'autorisation du conseil de surveillance ou d'administration, et c'est ce même conseil qui va ensuite fixer le montant et la durée de l'autorisation. Il s'agit donc d'une procédure relativement lourde, qui nécessite la réunion du conseil à chaque demande d'autorisation. Cette procédure entraîne par ailleurs une forte insécurité juridique pour nos sociétés en raison des incertitudes sur les montants autorisés. Cette situation est d'autant plus problématique que les sociétés sont aujourd'hui fréquemment amenées à apporter leur garantie à l'une de leurs filiales, en particulier pour des opérations conduites dans le cadre de marchés publics internationaux, qui requièrent parfois des capacités financières dont les filiales ne disposent pas. À l'aune de ces différents éléments, la proposition visant à autoriser l'octroi de la garantie par le conseil, sans limite de montant, sous la forme d'une garantie globale, permettra de sécuriser l'environnement juridique dans lequel évoluent les sociétés. Nous sommes donc face à une mesure certes technique, mais également pragmatique, dont on ne peut douter de l'utilité pour les entreprises. Mes chers collègues, le groupe Union Centriste, vous l'avez compris, votera en faveur de ce texte, dont les mesures répondent aux attentes et aux besoins des entreprises. Nous espérons que le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dont la simplification

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux à mon tour saluer l'initiative de Thani Mohamed Soilihi, ainsi que

qui résultent d'une complexité inutile, on va dans le bon sens ! Les mesures que vous proposez sont assurément positives. Je vais simplement mettre l'accent sur certaines d'entre elles. S'agissant des fonds de commerce, la mesure qui tend à supprimer les informations qui doivent être mentionnées par le cédant

même, l'idée d'encourager le recours au régime de la location-gérance des fonds de commerce en supprimant la condition selon laquelle le loueur doit avoir exploité le fonds pendant deux ans est nécessaire. Je regrette que l'Assemblée nationale se soit opposée à ces deux dispositions qui ont été présentées à la faveur d'autres textes. S'agissant maintenant des sociétés civiles, de l'article 10 qui permet la dématérialisation des formalités de cession de parts de société civile auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'instar de ce qui a été fait pour les SARL. Là encore, il aurait été archaïque de continuer à vivre dans un contexte où cette dématérialisation n'aurait pas été possible : ce n'est vraiment pas conforme aux objectifs qui sont les nôtres

S'agissant des sociétés anonymes, vous prévoyez la démission d'office du mandataire social placé lui aussi en tutelle ou curatelle.

de regrouper dans un document de référence unique l'ensemble des informations qu'elles sont légalement tenues de publier, comme le rapport de gestion du conseil, le rapport du président, les comptes annuels ou les données sociales et environnementales : que de papier !

la proposition que vous faites d'autoriser la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées va dans le bon sens. en outre favorable à cette autre disposition qui permet d'assouplir les périodes d'interdiction d'attribution aux salariés de stock-options ou d'actions gratuites pour favoriser l'actionnariat des salariés

des comptes aux associations et autres entités du secteur non marchand lorsque le total de leur bilan, leurs ressources et le nombre de leurs salariés sont inférieurs à des seuils fixés par décret. Que l'on puisse aider les associations est une bonne chose, et je crois que personne ne s'en plaindra. Mes chers collègues, je n'ai pas fait le compte exhaustif

Celle-ci s'appliquera fort longtemps, puisqu'il faut attendre 1807 pour que le code de commerce napoléonien voie le jour à la suite des faillites des fournisseurs aux armées, qui auraient pu entraîner la chute de la nouvelle Banque de France.

D'un point de vue historique, l'évolution du code de commerce a été laborieuse et la version de 1807 n'est qu'une pâle copie des ordonnances du XVII siècle. Le code de commerce de 1807 s'étoffera considérablement en deux cents ans : l'ordonnance du 18 septembre 2000 est venue codifier de multiples textes apparus hors du code,

Aujourd'hui toujours en vigueur, le nouveau code de commerce du 18 septembre 2000 ne cesse d'évoluer. En apparence, la codification et le commerce semblent former un couple bien difficile à unir pour longtemps l'une fige le droit, l'autre est en mouvement perpétuel. Oui, la rigidité du droit semble parfois bien incompatible avec le mouvement économique. Aussi, le droit du commerce ne supporte la codification que si celle-ci reste ouverte à toutes les évolutions. C'est pourquoi le processus de simplification du droit des entreprises est un chantier permanent, certes difficile, où de nouvelles initiatives doivent toujours être prises. Le but de ce processus est de clarifier, de rendre l'environnement juridique des entreprises davantage prévisible et d'alléger les formalités et démarches auxquelles elles sont soumises. Élaborée à la suite des travaux de notre collègue Thani Mohamed Soilihi- de nombreuses fois cité aujourd'hui -en sa qualité de rapporteur de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, la proposition de loi de soixante articles que nous examinons aujourd'hui est circonscrite pour l'essentiel au droit des sociétés et se situe dans le processus permanent de simplification de l'environnement juridique des entreprises.

La commission des lois a adopté soixante amendements sur la proposition de son rapporteur. Outre douze articles supprimés, car déjà satisfaits par d'autres textes, la commission a supprimé six articles dont la pertinence ne semblait pas avérée au regard de l'objectif de simplification. Elle a amélioré la rédaction de nombreux articles et a introduit neuf articles additionnels. Les principales mesures adoptées dans ce texte visent notamment à dématérialiser les formalités de publicité concernant la cession de parts de société civile, à permettre de régulariser la prorogation d'une société au-delà de son terme normal en cas d'oubli par les associés des formalités de prorogation, ou encore à dématérialiser les assemblées les assemblées générales des sociétés anonymes. Celles-ci tendent également à faciliter l'octroi par une société mère de sa garantie à ses filiales et à supprimer l'obligation de soumettre tous les trois générale une augmentation de capital réservée aux salariés. Elles clarifient en outre les règles d'attribution gratuite d'actions aux salariés. Enfin, elles simplifient les obligations de publicité incombant aux sociétés cotées par l'établissement d'un document unique et suppriment la solidarité fiscale dans le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce. À l'issue des travaux de la commission des lois, le texte renommé « proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés » regroupe cinquante mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous réjouissons de la permanence du processus de simplification du droit. La simplification et la modernisation de l'environnement juridique des entreprises contribuent à accroître leur compétitivité en facilitant et en sécurisant l'exercice de leurs activités.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans une économie mondialisée et concurrentielle, l'adaptation constante du droit des sociétés est un impératif, afin de doter nos entreprises des moyens juridiques de développer leurs activités et de garantir un environnement économique de confiance. C'est l'enseignement à tirer des travaux de l'économiste britannique Douglass North, récompensé par un prix Nobel pour ses recherches sur les institutions. En France, la matrice du droit des sociétés est définie par la loi du 24 juillet 1966, qui a bien été amenée à évoluer pour s'adapter aux mutations de l'économie. Plusieurs innovations ont ainsi utilement accompagné nos entreprises je pense en particulier au succès de l'ouverture du statut de société anonyme simplifiée- les SAS -à l'ensemble des entreprises par la loi du 12 juillet 1999. Lors du précédent quinquennat, de nombreuses dispositions ont été introduites dans la loi pour simplifier la vie de l'entreprise et relancer la croissance et l'activité. Nous les avons soutenues La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit directement dans l'esprit de ces précédents textes, puisqu'elle agrège le reste des mesures identifiées par notre collègue Thani Mohamed Soilihi lorsqu'il en était rapporteur qui n'y avaient pas été intégrées. Si nous sommes favorables à la plupart des dispositions de cette proposition de loi, nous sommes en revanche plus réservés sur le choix du véhicule législatif, alors que le Gouvernement a annoncé vouloir soumettre au Parlement un projet de loi intitulé « plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises »-

de ne pas faire obstacle au travail de notre collègue nous a donc conduits à retirer un certain nombre d'amendements. Nous considérons néanmoins que les circonstances de cet examen ne sont pas optimales. Comme je l'évoquais, plusieurs dispositions prévues à l'origine ont été introduites dans d'autres lois,

Ce calendrier particulièrement étendu dans le temps a contraint le rapporteur à déposer de nombreux amendements de coordination en séance. Leur examen réduira un peu plus nos débats sur le fond des dispositions proposées, par ailleurs très techniques. Nos réserves portent également sur la terminologie de la « simplification », qui devient l'alpha et l'oméga de l'initiative législative. Cette terminologie masque parfois le caractère « fourre-tout » de textes, dont on ne sait plus définir le sens ni la colonne vertébrale. cette proposition de loi aurait gagné en clarté en se limitant à l'adaptation du droit des sociétés anonymes au nouveau contexte économique, puisque ce sujet en est le coeur. De nombreuses ordonnances ont été prises en parallèle, comme les ordonnances ayant trait à la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés la simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence. Leur ratification, telle que proposée, aurait pour conséquence de rendre obsolètes d'autres dispositions, comme le rapporteur en a également pris acte. Depuis plusieurs années, le législateur veille à préserver la sécurité juridique des acteurs économiques et à garantir une relative stabilité du droit. Nous estimons que la multiplication de véhicules législatifs de simplification n'est pas de nature à permettre une bonne lisibilité des réformes, et s'éloigne de cet objectif de sécurité. Sur le fond, parmi la quarantaine d'articles restant d'actualité, plusieurs dispositions auraient mérité des discussions approfondies, afin de juger de leur impact. Je n'en citerai qu'une : la modification des règles de vote au sein des assemblées générales. Sur ce point, si une évolution de la prise en compte des abstentions par les actionnaires semble pertinente, celles-ci étant actuellement comptabilisées comme des votes négatifs, certains membres de mon groupe auraient souhaité que cette mesure s'accompagne d'une modification importante des règles de quorum des assemblées générales, afin de permettre aux actionnaires de s'adapter progressivement à la nouvelle donne. D'une façon générale, nous restons dans l'attente de débats approfondis sur les liens entre sociétés anonymes et économie réelle. Une récente étude publiée par et l'Institut de l'entreprise souligne les écarts de confiance des Français envers les entreprises, selon leur taille : 90 % d'opinions : 90 % d'opinions favorables pour les PME contre 44 % pour les grandes entreprises. Ces chiffres appellent à la réflexion ! Les grandes sociétés anonymes pâtissent encore trop souvent de la perception dégradante de nos concitoyens, qui les

En période de tarissement des capacités de financement, la popularisation du régime de la société anonyme devrait être davantage encouragée, y compris auprès des entreprises plus petites.

et les entreprises de taille intermédiaire à compter au moins 40 % de femmes dans leur conseil d'administration, ce qui n'est pas encore le cas. Malgré ces quelques réserves, le groupe du RDSE portera sur ce texte

des mentions obligatoires devant être portées sur l'acte de cession, en raison de leur caractère aujourd'hui inadapté et incomplet. Je voudrais remercier Pierre-Yves Collombat d'avoir bien voulu retirer son amendement. Effectivement, la suppression complète ne s'impose

Cet amendement de précision vise à actualiser la proposition de loi, en reprenant une rédaction améliorée, adoptée en son temps par le Sénat dans le cadre de la loi Sapin II. Il porte sur le mécanisme de régularisation, sur autorisation judiciaire, de la prorogation d'une société.

sous-amendement

Le sous-amendement n° 16 tend à supprimer des mesures de simplification des obligations comptables et des obligations de publication applicables aux petites entreprises, pourtant permises par le droit européen.

dans le cadre de la loi Sapin II. Cette actualisation concerne les modalités de remplacement du gérant d'une société à responsabilité limitée en cas de vacance ou de placement en tutelle.

Cet amendement de précision vise à reprendre la rédaction adoptée en son temps par le Sénat, dans le cadre de la loi Sapin II. Il porte sur l'assouplissement des conditions d'octroi de la garantie d'une société mère à ses filiales contrôlées, par le conseil ou par le directeur général de la société. Nous y avons Nous y avons déjà fait allusion dans le cadre de la discussion générale.

Comme cela vient d'être dit, cet amendement vise à actualiser la proposition de loi pour tenir compte de modifications introduites dans le code de commerce par l'ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés. La suppression de l'article 19 s'impose.

8 est retiré.

ainsi libellé : La parole est à M. le rapporteur. Il s'agit simplement d'un amendement de correction d'une erreur matérielle issue de l'ordonnance du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information

L'article 23 tend à permettre la dématérialisation des assemblées générales dans les sociétés non cotées. S'il est effectivement satisfait par une disposition prise par ordonnance en 2017, cette disposition soulève une difficulté, que l'amendement suivant de M. Thani Mohamed Soilihi vise utilement à résoudre.

Ce droit d'opposition aurait eu davantage de sens si la réunion dématérialisée avait été prévue comme une faculté par la loi. C'était d'ailleurs l'architecture initiale de la proposition de loi, que nous avons modifiée sur ce point en commission. Dans ces conditions,

: La parole est à M. le rapporteur. Cet amendement de coordination vise donc à tenir compte des modifications introduites dans le code de commerce par l'ordonnance du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés.

on le sait bien, une telle résolution est systématiquement rejetée par les assemblées générales, ce qui, vous en conviendrez, monsieur Collombat, n'est pas un très bon signal pour l'actionnariat salarié ... En fait, le conseil d'administration doit présenter une résolution dont il demande ensuite le rejet ! C'est incompréhensible, en particulier par les investisseurs étrangers, mais aussi, comme j'ai eu l'occasion de le constater moi-même, par bon nombre d'associés, qui ne sont pas au fait des arcanes de la loi et qui ne comprennent pas comment l'on peut présenter une résolution dont on demande le rejet juste après. J'ajoute que la proposition de loi conserve l'obligation de présenter à l'assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés dès lors qu'on lui présente une augmentation de capital classique. Nous aurions pu aller plus loin,

Ce qui est bien avec Pierre-Yves Collombat, c'est que c'est un visionnaire ! Cet amendement se situe en effet dans la continuité du débat sur l'article 27. Il est contraire à la position de la commission. Aujourd'hui, lorsqu'on ne soumet pas à l'assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés parallèlement à toute augmentation de capital classique, cette augmentation de capital peut être annulée, ce qui est un risque juridique important. Par cet article, il est simplement de remplacer cette sanction de nullité par une injonction de faire, plus efficace qu'une nullité, et qui permettrait, par exemple, à un salarié d'exiger l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une augmentation de capital réservée aux salariés,

depuis 2012, plusieurs sanctions pénales relatives aux infractions au droit des sociétés ont été supprimées. Plusieurs dispositions de la proposition de loi, figurant aux articles 25 et suivants, visaient à affaiblir les conséquences de manquements à certaines règles définies par ce droit. Cela ne nous semble pas être une évolution satisfaisante, dès lors qu'elle reviendrait à transformer ces règles en droit mou, à valeur indicative plutôt que dissuasive. Le rapporteur a déjà procédé à des modifications, afin d'atténuer les transformations proposées par le présent texte. Dans son rapport, publié en 2016, il a, par exemple, justifié la suppression de l'article 32, en considérant qu'il était « nécessaire de conserver un niveau de sanction plus élevé, afin d'éviter tout risque d'omission délibérée par le conseil de la formalité de publicité de l'opération. » Un raisonnement identique n'est-il pas applicable à la disposition qu'il propose à l'article 29 ?

la sanction de suspension des droits de vote pour les actions irrégulièrement émises est grave, source de sérieuse insécurité juridique pour les décisions prises par ignorance sur la base de ces droits de vote.

Le Gouvernement n'est pas favorable à la suppression de toute sanction en cas de méconnaissance des règles applicables en matière d'augmentation de capital. Cela rejoint la préoccupation de M. Requier. Simplement, il faut que la sanction soit proportionnelle.

l'avis du Gouvernement ? Certes, c'est un amendement de coordination, mais, malgré tout, raccourcir la période de calcul du prix de souscription

Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination concernant l'assouplissement des périodes d'interdiction de cession des actions gratuites attribuées aux salariés et la clarification du champ des personnes concernées par cette interdiction. Cet amendement tend également à assurer une mise en conformité avec le droit européen, fixe une période d'interdiction de trente jours calendaires pour les dirigeants des sociétés concernées. Dans un souci de simplification, il retient ce même délai pour les dirigeants comme pour les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée.

émet un avis éminemment favorable ! Cet amendement apporte plusieurs mesures utiles de simplification ou de souplesse dans les règles de rachat par une société non cotée de ses propres actions, sans remettre en cause les principes de ce dispositif ni les garanties pour les actionnaires.

portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés. Quel est l'avis du Gouvernement ? J'insiste

est à M. le rapporteur. Le présent amendement vise à actualiser la proposition de loi, pour tenir compte de l'adoption d'une partie de cette disposition dans le cadre de l'ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés. Il s'agissait de permettre de modifier les clauses d'agrément d'un nouvel associé à la majorité plutôt qu'à l'unanimité des associés. La même modification demeure dans le texte pour ce qui concerne les clauses de retrait d'un associé.

mais également les experts-comptables.

de la proposition de loi concernant l'obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant, le risque de défaillance ou d'empêchement du commissaire aux comptes titulaire étant quasi nul du fait de l'exercice en société aujourd'hui de la très grande majorité des commissaires aux comptes.

partisan de la simplification de la vie des entreprises, votera bien entendu ce texte. Il remercie M. le ministre d'aller encore plus loin dans le pacte pour améliorer la situation de celles-ci dans notre pays.

qu'aller à un train de sénateur voulait dire aller plus vite que la lumière, ce qui n'est pas ma compréhension habituelle de cette expression ! C'est la preuve que cette assemblée est capable d'adopter rapidement des textes quand ceux-ci vont dans le sens de l'intérêt général.

Merci,